Madame la présidente,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

Pour éviter les dégradations et pillages, nombre d'entre eux ont préféré baisser le rideau, se privant ainsi de ce chiffre d'affaires dont ils ont tant besoin. D'autres, pourtant situés à l'écart des zones de manifestations, ont constaté une baisse de fréquentation.

Dans 93 % des cas, il s'agissait de petites et moyennes entreprises. Il est donc urgent que cette situation cesse. Or de nouveaux mouvements de grève sont annoncés pour jeudi prochain, pour manifester contre la réforme des retraites voulue par le Gouvernement, qui pourraient avoir des conséquences négatives, à leur tour, sur nos commerces. Il est bon de rappeler que les commerçants ne sont pas responsables des tensions qui se manifestent dans la rue. Eux aussi sont excédés par les taxes et les impôts. Eux aussi sont victimes de réglementations trop strictes qui les étouffent. Il est important que les participants aux manifestations passées ou à venir comprennent que la disparition programmée de ces milliers de commerçants

et à l'élaboration de l'opération nationale « revitalisation et animation des commerces » pour les centres-villes. Le 16 mai 2019, nous sommes venus en appui de trente-cinq collectivités, dans onze régions, en cofinançant à hauteur de près de 6 millions d'euros leurs projets d'animation, d'attractivité et de communication commerciales.

touchées par la contractualisation avec l'État, ainsi que par les contraintes qui en résultent, ce qui a pour effet de limiter leurs actions, notamment dans les zones sensibles. En effet, parmi les 322 collectivités qui ont contractualisé avec l'État et qui doivent respecter un taux de croissance de 1,2 % en moyenne par an de leurs dépenses de fonctionnement, nombreuses sont celles qui portent de longue date des politiques volontaristes de coopération décentralisée, et pour certaines en zones très sensibles. Or l'administration oblige actuellement les collectivités à intégrer dans leur budget principal les recettes et les dépenses de coopération, alors même que, si les collectivités sont engagées sur leurs propres participations financières, elles servent souvent de simple « boîte à lettres » entre les financeurs extérieurs et les acteurs implantés localement. À ce jour, les collectivités peuvent se trouver en difficulté et s'interrogent sur leur capacité à poursuivre certaines de leurs actions. Cela est d'autant plus lourd de conséquences quand il s'agit de territoires sensibles, j'y insiste,

zones difficiles, voire dangereuses, et où l'appui à des coopérations installées depuis de nombreuses années serait particulièrement utile. Il apparaît donc nécessaire d'obtenir une adaptation de la réglementation pour que les financements obtenus de l'extérieur de la collectivité, et pour lesquels la collectivité n'est qu'un intermédiaire, ne soient pas pris en compte dans la limite imposée dans le cadre de la contractualisation. du débat sur le projet de budget de l'aide au développement, a donné un certain nombre d'assurances. Pouvez-vous, monsieur le secrétaire d'État, nous confirmer les engagements du Gouvernement et nous dire quelles mesures pourraient être prises rapidement pour régler cette situation délicate ?

précise les conditions dans lesquelles l'État propose à 322 collectivités en France de signer un contrat de maîtrise de l'augmentation des dépenses de fonctionnement. Ce point est important car, sur ces 322 collectivités, 230 environ ont accepté de signer et de s'engager à maîtriser l'augmentation de ces dépenses. Je parle bien de « maîtriser » cette augmentation car, vous l'avez rappelé, c'est non pas une diminution des dépenses de fonctionnement qui est attendue, mais une maîtrise de leur augmentation à hauteur de 1,2 % par an pendant trois ans, et de manière cumulative.

que le montant total affecté aux dotations de fonctionnement, autour de 27 milliards d'euros, est maintenu en 2020 pour la troisième année consécutive après, vous le savez, quatre années de baisse des dotations pour un montant total de 11 milliards d'euros.

L'objectif est de mesurer la maîtrise des dépenses et l'amélioration de la capacité de financement sur un périmètre identique. À nos yeux, l'évolution des dépenses exposées par une collectivité au titre de la coopération décentralisée ne relève ni d'un transfert de compétences ni d'un élément exceptionnel susceptible de fausser la comparaison entre deux exercices. En effet, pour les dépenses qui étaient déjà inscrites en 2017, cela est pris en compte dans la référence de départ. La participation volontaire d'une collectivité au financement d'une action qui bénéficie par ailleurs de cofinancements à des titres divers ne peut être considérée, aux termes de l'article 29 de la loi de programmation, comme relevant d'une dépense exceptionnelle. Ces actions qui participent des modalités classiques d'intervention des collectivités

sur les contrats de Cahors et de voir comment en améliorer le fonctionnement. D'ici là, les dépenses que vous citez sont prises en compte dans le périmètre, mais, je le répète, il convient d'avoir en tête que, pour toutes les collectivités qui menaient déjà ses actions 2017, cela était déjà prévu dans le périmètre de départ. L'évolution tient donc compte, aussi, de ce qui existait préalablement.

Un département rural comme le mien, la Nièvre, a ainsi perdu 74 postes en équivalents temps plein (ETP) depuis 2015. À l'appui de cette réorganisation, le ministère de l'action et des comptes publics invoque le principe de « déconcentration de proximité ». Ce principe est censé redistribuer l'implantation du réseau de la DGFiP, à l'échelle nationale comme à l'échelle locale, des métropoles et chefs-lieux de département. Au-delà des problématiques de répartition territoriale, se pose la question des moyens humains affectés aux services décentralisés et centraux, notamment dans le contexte de la réforme du prélèvement à la source. À quel niveau sera fixé le socle minimal

Nous installerons également sur le territoire, soit dans des bâtiments occupés par les finances publiques, soit en partenariat avec le réseau France Services ou les intercommunalités, 1 200 conseillers aux décideurs locaux, qui sont des agents des finances publiques spécifiquement chargés du conseil aux élus, sur l'ensemble du territoire, intercommunalité par intercommunalité.

Les initiatives innovantes en faveur de l'emploi sont encouragées par le département. C'est dans ce cadre que la commune de Pontchâteau s'est engagée dans le dispositif « Territoires zéro chômeur de longue durée », dont le principe de l'expérimentation pour dix territoires venait d'être rendu possible par la loi. Si sa candidature n'a pas été retenue en 2016, le territoire s'est néanmoins fortement investi et organisé dans la perspective d'une deuxième étape d'expérimentation. Ainsi, depuis plus de deux ans, tous les acteurs locaux ont été inclus dans la démarche et réunis plusieurs fois en comité de pilotage local. Une dynamique territoriale nouvelle s'est enclenchée avec enthousiasme. La préfiguration de cette expérimentation soulève beaucoup d'espoirs sur le territoire de Pontchâteau, qui compte 410 chômeurs de longue durée. durée. Le Président de la République ayant mentionné lui-même le dispositif « Territoires zéro chômeur de longue durée » au moment des annonces sur la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, le 13 septembre 2018, les acteurs locaux s'attendaient à une accélération du calendrier, permettant enfin aux dizaines de personnes mobilisées de retrouver le chemin de l'emploi durable. Dès lors, l'absence de perspectives à la suite des annonces présidentielles suscite beaucoup d'incompréhension. Pouvez-vous m'indiquer quelles seront les prochaines initiatives du Gouvernement

chômage. L'expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée, prévue par la loi du 29 février 2016, a été lancée de manière opérationnelle en janvier 2017. Nous en sommes donc à trois années de mise en oeuvre. oeuvre. Depuis 2017, douze entreprises à but d'emploi ont été créées sur les dix territoires retenus après appel à projet, et 900 personnes privées d'emploi ont pu être recrutées, dont 750 sont actuellement salariées. Nous pouvons nous féliciter de ces chiffres. Je peux vous assurer, à ce titre, du plein soutien du ministère du travail à cette démarche expérimentale. En 2020, seront financés 1 000 ETP supplémentaires par rapport à la prévision de réalisation pour 2019, et ce en cohérence avec la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté.

expérimentation est intéressante, car elle permet de tester des modalités innovantes de lutte contre le chômage de longue durée. Parmi ces innovations figurent notamment l'approche territoriale et la mobilisation des élus locaux, qui constituent une condition de réussite du projet.

C'est dans ce sens que la ministre du travail a réuni, lundi 25 novembre dernier, M. Laurent Grandguillaume, qui s'occupe de l'association portant cette expérimentation, le comité scientifique qui a remis son évaluation intermédiaire, ainsi que les inspecteurs de l'inspection générale des affaires sociales

Priou, pour la réplique. « Le chômage n'est pas une fatalité », déclarent souvent les candidats aux élections, quels que soient les échelons territoriaux d'ailleurs. Certes ! Mais n'attendons pas les mauvais cycles économiques pour enclencher une dynamique vertueuse sur les territoires qui en prennent l'initiative.

ministre de l'intérieur. Monsieur le secrétaire d'État, je souhaite attirer votre attention sur la mise en péril du budget de la commune de La Mure, en Isère, dans le cadre de l'exécution du bail de sous-location de la gendarmerie, que la commune a fait construire sur son territoire. Ces difficultés tiennent au fait que le montant des loyers versés par la commune n'est pas intégralement couvert, tant s'en faut, par celui des loyers que l'État lui verse pour l'occupation de la gendarmerie. La différence, selon la nouvelle révision triennale, s'élèverait à 150 000 euros par an, ce qui représente une somme insupportable pour le budget de la commune.

Dans la première réévaluation du loyer par la DGFiP, c'est bien cette évaluation des loyers selon l'ICC qui a été établie. Or il se trouve qu'un autre contrat de sous-location, différent de celui qui a été soumis aux élus, précise que la révision se fait selon la valeur locative. Cette disposition « valeur locative » est la plus dommageable à la commune et la mettrait en difficulté avec ce delta annuel de 150 000 euros. Deuxièmement, la commune a confié la construction de cette gendarmerie à la société Auxifip par le biais d'un bail emphytéotique. Or, non seulement les loyers dus par la commune à cette société n'ont pas été arrêtés au regard des loyers que la commune devait percevoir et perçoit aujourd'hui de l'État, mais le plan de financement d'Auxifip repose sur un emprunt à taux fixe de 4,75 %.

Il semblerait en effet qu'un groupe interministériel soit créé pour permettre à plusieurs communes de se fédérer et de peser face à Auxifip, afin de renégocier des taux de crédit acceptables. Par ailleurs, et dans cette attente, il est impératif de poursuivre

j'entends votre inquiétude. En effet, certains montages financiers de baux emphytéotiques ont fait apparaître une décorrélation, parfois significative, entre le loyer versé par l'État à la collectivité et le loyer que la collectivité acquitte au constructeur ou au bailleur. Je vous confirme qu'une vingtaine de communes ayant conclu ce type de montage ont fait état de leurs difficultés financières à l'occasion du renouvellement de certains baux. La raison de ce décalage est la suivante : d'une part, la collectivité négocie avec le constructeur-bailleur un plan de financement adossé aux taux d'emprunts pratiqués sur les marchés financiers au jour de la signature du contrat ; d'autre part, le loyer versé par l'État à la collectivité doit correspondre à un loyer conforme à un marché locatif local. Il est d'ailleurs prévu, dans chaque contrat de bail de l'État, de plafonner l'actualisation du loyer en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction. Il convient de rappeler que l'État n'a pas vocation à devenir propriétaire de la caserne. En effet, à l'issue du bail entre la collectivité et le constructeur, l'immeuble revient en pleine propriété à la collectivité. Nous sommes donc face à deux contrats qui ne peuvent être assimilés : d'une part, celui de la collectivité, qui a vocation à devenir propriétaire des lieux ; d'autre part, celui de l'État, qui n'est que l'occupant pour une durée limitée. Pour autant et malgré cette nécessaire distinction, il convient de prendre en compte les difficultés financières que rencontrent certaines collectivités et que vous avez rappelées, madame la sénatrice. C'est pourquoi un groupe de travail a été installé le 16 octobre dernier. Il est chargé de mettre en place le plus rapidement possible un dispositif concret d'accompagnement dans la renégociation renégociation des clauses financières des contrats passés avec les constructeurs-bailleurs. Dans l'attente de l'élaboration d'une stratégie globale de rééquilibrage, les difficultés des communes sont examinées avec la plus grande attention pour que, dans chaque situation évoquée, des solutions soient recherchées et qu'un accompagnement individualisé puisse être mis en place. La commune de La Mure doit pouvoir bénéficier de cet accompagnement personnalisé en se rapprochant des services locaux du domaine de l'État. La parole

Le mode d'élection des conseillers généraux, rebaptisés « départementaux », a été modifié avant le renouvellement de 2015. Or le nouveau système, qui comprend des binômes homme-femme, présente de nombreux inconvénients. D'une part, il arrive souvent qu'au sein d'un binôme les rapports soient très conflictuels. D'autre part, le redécoupage des cantons a été arbitraire et ceux-ci n'ont plus aucune cohérence territoriale. Enfin, ce mode de scrutin doublement majoritaire est encore plus incompatible que le précédent avec un minimum de représentation du pluralisme politique. Afin de remédier à ces problèmes tout en garantissant des majorités de gestion, ne serait-il pas possible d'instaurer pour les élections départementales un mode de scrutin proportionnel avec prime majoritaire ? Cela pourrait ensuite faciliter des rapprochements conduisant, à terme, au rétablissement du conseiller territorial, exerçant à la fois les fonctions de conseiller départemental et celles de conseiller régional.

calendrier électoral a modifié le mode de scrutin pour l'élection des conseillers départementaux en instaurant un scrutin binominal paritaire majoritaire à deux tours, afin, d'une part, de conserver le lien étroit entre l'élu et son territoire, et, d'autre part, de favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux fonctions électives. La part des femmes siégeant au sein des conseils départementaux est ainsi passée de 13,5 13,5 %, en 2013, à 50 %, lors du renouvellement général de mars 2015. Le scrutin binominal ne lie les candidats qu'au moment de leur élection. Une fois élu, chacun des membres du binôme exerce son mandat de façon indépendante. Une mésentente n'affecte donc pas le fonctionnement du conseil départemental. Le redécoupage de l'ensemble des cantons a obéi à des critères démographiques, seuls garants de l'égalité de la représentation des citoyens. Les quelques dérogations au respect de l'équilibre démographique entre les cantons d'un même département ont été justifiées par un motif d'intérêt général, en respectant la jurisprudence du Conseil constitutionnel et du Conseil d'État. Ce redécoupage n'a nullement revêtu le moindre caractère arbitraire ; du reste, plus de 2 600 recours ont contester les décrets de 2014 délimitant les nouveaux cantons et aucun d'eux n'a prospéré. Vous souhaitez savoir si les conseillers départementaux pourraient être élus au scrutin proportionnel avec une prime majoritaire. Après de nombreuses discussions, en 2013, le choix de la lisibilité du mode de scrutin pour l'ensemble des électeurs l'a emporté, au travers du maintien d'un mode de scrutin majoritaire dans le cadre d'un canton.

de vue de la gouvernance, une élection des conseillers territoriaux à la proportionnelle avec attribution d'une prime majoritaire à l'échelle départementale ne garantirait nullement l'émergence d'une majorité au conseil régional, ce qui ferait courir un risque important de blocage institutionnel. Enfin et surtout, pour respecter l'égalité démographique entre les départements au sein de chaque région, désormais plus vaste, le nombre de conseillers territoriaux à élire pourrait rendre certaines assemblées pléthoriques. Pour ces raisons, le Gouvernement ne souhaite pas engager de réflexion relative au rétablissement du conseiller territorial. La parole

une dose de proportionnelle pour l'élection des députés, en soulignant que le mode de scrutin uninominal majoritaire était une distorsion inacceptable par rapport à la légitime représentation démocratique des suffrages.

sur la cohérence des découpages des cantons. Vous le savez très bien, le Conseil d'État ne s'est prononcé que sur l'équilibre démographique

pour satisfaire des arbitrages politiques, ce qui est de bonne guerre- le gouvernement de M. Sarkozy avait fait pire au moment des législatives -, mais il n'y a plus aucune cohérence territoriale des cantons,

(SIV). C'est aujourd'hui l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) qui assure la maîtrise d'oeuvre du SIV, en lien avec plusieurs services du ministère de l'intérieur. Le fonctionnement de ce système est satisfaisant dès lors que l'on reste dans un cadre simple, c'est-à-dire soit pour l'immatriculation d'un véhicule livré en concession et non par un mandataire, soit pour l'immatriculation d'un véhicule d'occasion déjà immatriculé en France, sans modification de ses caractéristiques. Toutefois, dans le cas d'importations ou de modifications, le système n'est pas adapté. En effet, en cas de problème, il est impossible de joindre le moindre interlocuteur. Seul un numéro de téléphone permet de contacter un service, basé à Charleville-Mézières, composé d'un personnel, certes de bonne volonté, mais qui n'a pas la capacité de donner suite aux demandes formulées. Ce service ne peut qu'envoyer une alerte au centre de traitement. Il est donc impossible de joindre ou de transmettre un complément d'information ou un document, si le gestionnaire du dossier ne recontacte pas le demandeur par message, le site internet de l'ANTS. Certains messages laissent d'ailleurs à penser que le personnel chargé de traiter les dossiers ne maîtrise pas les spécificités de chaque cas et manque significativement d'expérience, notamment sur les points particuliers liés à la fiscalité ou à des éléments techniques. Enfin, le site internet présente des dysfonctionnements qui n'ont jamais été corrigés ; je pense ici à des messages d'information envoyés en plus de dix exemplaires ou à des dossiers en cours d'analyse alors qu'une seconde demande a déjà été traitée. Monsieur le secrétaire d'État, quelles mesures seront mises en place pour que l'ANTS dispose d'un outil informatique fonctionnel et pour qu'une réelle assistance téléphonique puisse être créée, afin de garantir et de simplifier les démarches menées par les utilisateurs, plus particulièrement pour les professionnels ?

Lorsque l'une de ces opérations nécessite la production d'un certificat d'immatriculation, celui-ci est envoyé au domicile de l'usager en moins de trois jours, en France métropolitaine. Les enquêtes de satisfaction pour ces opérations montrent que plus de 70 % des usagers sont satisfaits. 5 % des opérations sont plus complexes et nécessitent des contrôles plus poussés. Aujourd'hui, l'administration instruit ces opérations dans un délai moyen de quinze jours. Les dossiers transmis par les usagers sont parfois incomplets, ce qui augmente ce délai. Lorsque les procédures se faisaient aux guichets des préfectures, il en allait de même et il arrivait régulièrement que l'usager doive revenir pour produire une pièce manquante. Cela dit, des améliorations sont toujours possibles. Ainsi, depuis 2018, 16 modifications ont été apportées au logiciel pour améliorer l'ergonomie des téléprocédures et simplifier le parcours de l'utilisateur. Par ailleurs, l'accompagnement des usagers a été renforcé, avec les points d'accueil numérique, en préfecture et en sous-préfecture, mais surtout avec le renforcement du « centre de contact citoyens » de l'ANTS. Ce centre de contact peut être joint par téléphone, par courriel ou sur les réseaux sociaux, 6 jours sur 7. De 60, en 2017, nous sommes passés à près de 300 téléconseillers, qui répondent en moins de 48 heures aux messages. Au téléphone, le temps d'attente est inférieur à 5 minutes. Enfin, un parcours guidé a été mis en place sur le portail de l'ANTS, pour aider les usagers à réaliser les démarches relatives à l'immatriculation des véhicules les plus complexes, et l'ANTS travaille à la refonte complète de son site internet afin de le rendre plus pratique, accessible et clair. l'échelon ministériel, l'instance nationale d'écoute « usagers » et ses deux groupes de travail se réunissent régulièrement. De nombreux moyens de mesure de la satisfaction ont été développés. Les résultats de l'action du ministère sont visibles : l'ANTS a ainsi été élue service client de l'année 2020,

de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes), créée en 2002, a pour mission d'observer et d'analyser le phénomène des dérives sectaires, d'informer le public sur les risques que celles-ci représentent et de coordonner l'action préventive et répressive des pouvoirs publics.

La rationalisation des services de celui-ci ne doit pas conduire à la suppression ou à la restructuration de cette mission au sein du Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation. le sujet des dérives sectaires ne saurait être soluble dans la problématique de la prévention de la radicalisation, sauf à vouloir faire un cadeau aux groupes sectaires Prendre une décision en ce sens reviendrait à méconnaître totalement la dangerosité du phénomène sectaire, le nombre de ses victimes ainsi que l'efficacité de la structure interministérielle. Enfin, les personnes radicalisées ont un profil et un parcours totalement différents de ceux des personnes sous l'emprise d'une secte ; ils n'ont rien de commun. J'ai dirigé pendant vingt-cinq ans les études des étudiants de l'Institut d'études judiciaires de Lille II. Sur ma demande, la présidente départementale du Centre national d'accompagnement familial face à l'emprise sectaire Mme Charline Delporte, qui m'avait été présentée par M. le préfet, faisait part aux étudiants des violences, visibles ou non, subies par les enfants placés sous l'emprise de mouvements sectaires, afin de sensibiliser les futurs avocats et magistrats à ces problèmes.

avoir le sentiment que le Gouvernement diminue sa vigilance et laisse tomber la lutte contre les dérives sectaires en supprimant un outil que le monde entier nous envie. La parole est

connaissons, comme vous, l'importance des sujets liés à la prévention et à la lutte contre les dérives sectaires, sous toutes leurs formes et dans les différents secteurs de la vie sociale au sein desquels ces dérives peuvent aujourd'hui se manifester. J'ai déjà eu l'occasion de le rappeler, en répondant ici même au Gouvernement, ces dérives prennent des formes très évolutives et nécessitent un suivi le plus fin possible. Une part de l'activité de la Miviludes pose aujourd'hui des questions de synergie et de partage de compétences avec d'autres organismes, qui n'existaient pas au moment de la création de cette comme, effectivement, le secrétariat général du Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation. De plus, la Cour des comptes a formulé, en 2017, plusieurs observations sur l'organisation et le fonctionnement de la Miviludes, en évoquant l'option de son rattachement au ministère de l'intérieur. D'ailleurs, il est de bonne administration que l'action publique relève des ministères ; cela permet au Premier ministre et à ses services de se concentrer sur leur rôle d'impulsion, de coordination et d'arbitrage. C'est dans ce contexte que le Gouvernement a décidé de rattacher la Miviludes au ministère de l'intérieur, où elle pourra exercer ses missions en pleine articulation avec les missions exercées au titre de la lutte contre les nouvelles formes de radicalité et certains phénomènes d'emprise. Toutefois, je tiens à vous rassurer, madame la sénatrice, cette nouvelle organisation ne

d'action publique contre les dérives sectaires, et nous continuerons donc naturellement à y apporter les moyens nécessaires ; d'autre part, nous veillerons à ce que la nouvelle organisation préserve la bonne prise en compte de la spécificité des phénomènes sectaires. Bien évidemment, nous ne réduisons pas la question des dérives sectaires à la seule problématique de la radicalisation djihadiste ; que les choses soient dites clairement. Les missions de la Miviludes n'ont pas vocation à être dissoutes dans celles

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, le 7 octobre dernier, le directeur de la maison d'arrêt de Fontenay-le-Comte, en Vendée, faisait l'objet d'une violente agression de la part d'un détenu. Les faits sont d'une extrême gravité et soulignent un véritable problème de sécurité pour le personnel pénitentiaire, qui est amené à faire face à une surpopulation carcérale de plus en plus inquiétante dans les deux prisons vendéennes.

Je souhaite donc savoir si le Gouvernement compte tenir ses engagements sur ce montant, pour quels projets et pour quelle date de mise en oeuvre. Je souhaite également connaître les dispositions rapides qu'il entend prendre s'agissant de la situation de surpopulation carcérale des prisons vendéennes et de la sécurité du personnel pénitentiaire en général.

carcérale importante. Le 2 décembre 2019, le taux d'occupation de l'établissement s'élevait à 182 % : 71 détenus y étaient hébergés pour une capacité de 39 places. Des couchages supplémentaires ont été mis en place dans les cellules pour faire face à cette situation. Un suivi quotidien des effectifs et une politique de transfèrement de certains détenus condamnés, lorsque cela est possible, sont mis en place par l'administration pénitentiaire pour tenter de réguler les effectifs. Le 7 octobre dernier, le chef d'établissement de la structure a été victime d'une agression par un détenu du quartier disciplinaire, qui s'est traduite par une interruption temporaire de travail d'un jour. L'agresseur faisait l'objet d'une évaluation au regard d'éléments de radicalisation ainsi que d'un suivi régulier en raison d'un comportement notoirement violent. Dès le 8 octobre, ce détenu a été transféré dans un autre établissement. Au-delà de ce cas spécifique, le ministère de la justice a augmenté le budget consacré à la sécurité des établissements pénitentiaires et de son personnel ; ainsi, 58,1 millions d'euros sont inscrits au titre du projet de loi de finances pour 2020, soit une hausse de 16 % par rapport à 2019. 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice permet désormais d'affecter, au sein de quartiers spécifiques, comme des unités pour détenus violents ou des quartiers de prise en charge de la radicalisation, des détenus dont le comportement porte atteinte à la sécurité publique ou au bon ordre de l'établissement. Dans ce type de quartiers, les personnes détenues bénéficient d'un programme adapté de prise en charge et sont soumises à un régime de détention impliquant notamment des mesures de sécurité renforcée. L'objectif que nous visons est d'évaluer chaque détenu présentant des signes de violence ou de radicalisation, afin de décider d'une prise en charge pluridisciplinaire adaptée, en fonction du danger qu'il représente et du niveau de sa radicalité. Cette prise en charge peut se faire dans les quartiers d'isolement, dans les unités spécifiques que je viens d'évoquer ou en détention classique selon des modalités adaptées. particulier, les programmes de prévention de la radicalisation violente ont été généralisés. Ces programmes, d'une durée de trois à cinq mois, comportent des séances collectives et des entretiens individuels réguliers. Le déploiement progressif des binômes de soutien, actuellement au nombre de 90, composés d'un psychologue et d'un éducateur, a également permis de renforcer la capacité de l'administration pénitentiaire à prendre en charge les personnes radicalisées placées sous main de justice. Enfin, un plan de formation spécifique portant sur ces thématiques a été conçu à l'attention de l'ensemble du personnel de l'administration pénitentiaire, en priorité au bénéfice des professionnels prenant spécifiquement en charge des détenus violents ou présentant des signes

critique de l'établissement pénitentiaire. La semaine dernière, on comptabilisait 384 détenus hommes pour 222 places, réparties en 205 cellules, soit un taux Selon l'Observatoire international des prisons, la surpopulation carcérale à Caen est chronique depuis les années 1990, et le quartier des hommes présente, quasiment en permanence depuis dix ans, un taux d'occupation On peut le dire, les conditions de détention sont très difficiles. La prison actuelle date de 1904 ; certes, elle a évolué, mais- c'est une évidence -elle est d'un autre temps. Dans ce contexte tendu, une part très minoritaire du public hébergé bénéficie d'un encellulement individuel. Les détenus sont souvent trois, parfois quatre, nous dit-on, dans des cellules de 9 mètres carrés. Cette promiscuité augmente les tensions ; elle est source de violences. Cela a également des conséquences négatives sur le travail des conseillers en insertion et sur l'accès aux soins. On compte un peu plus de 80 surveillants pénitentiaires au quotidien, pour s'occuper des détenus de la maison d'arrêt, ce qui serait suffisant si le taux d'occupation était respecté ; mais ce n'est pas le cas. Difficile de protéger et de se protéger dans ces conditions. C'est un travail ardu qui demande une plus grande vigilance encore que dans des conditions dites « normales ». Les incidents sont nombreux, ils impliquent des sanctions disciplinaires et donc nuisent à l'obtention d'un aménagement de peine. Tout cela favorise la récidive, non la réinsertion. En 2022, une nouvelle maison d'arrêt verra le jour à Caen ; cela doit apporter une solution, mais, dans ces conditions, attendre trois années de plus est impossible. D'ici là, il faut agir. Monsieur le secrétaire d'État, quelles solutions proposez-vous, en attendant 2022, pour que cette situation ne perdure pas et que soient traitées la question de ces

Toutefois, l'établissement ne compte aucun matelas au sol ; des lits superposés ont été installés lorsque la superficie des cellules le permettait. Par ailleurs, même si l'on ne peut s'en satisfaire, seulement 2 % de la population pénale de l'établissement est hébergée dans des cellules de cinq places. Si les conditions de détention demeurent difficiles au sein de cette maison d'arrêt, il est à noter que 80 % des détenus sont affectés dans une cellule double ou individuelle. Le taux d'encellulement individuel de l'établissement est, au 2 décembre 2019, de 12,8 %. Bien qu'insuffisant, ce taux est en augmentation par rapport à celui du 1 octobre 2017, date à laquelle il s'élevait à 10,5 %. Afin de réguler le taux d'occupation de la maison d'arrêt, des détenus condamnés à de courtes peines ou dont le reliquat de peine est inférieur à deux ans ont été transférés, sur leur demande, vers des centres de détention. Ce suivi quotidien des effectifs et cette politique de transfèrement, lorsqu'elle est possible, seront maintenus. Si la maison d'arrêt de Caen connaît un taux de surpopulation à l'image d'autres maisons d'arrêt métropolitaines et ultramarines, des travaux y sont toutefois régulièrement réalisés afin d'améliorer les conditions de détention en 2016, les menuiseries extérieures et les sanitaires des promenades ont été rénovés ; en 2018, la chaudière du quartier des hommes a été remplacée et des travaux d'étanchéité de la toiture ont été réalisés en 2019, les cellules du quartier disciplinaire ont été remises à neuf, achevant ainsi le plan de rénovation de l'ensemble des cellules de l'établissement, commencé en 2015. je vous le confirme, la construction du nouveau centre pénitentiaire de Caen, d'une capacité de 551 places et d'un coût de 115 millions d'euros, commencera au troisième semestre 2020, pour s'achever en fin d'année 2022. Enfin, une structure d'accompagnement à la sortie, d'une capacité de 90 places, verra également le jour à Caen. Les travaux commenceront au cours de l'année 2020, pour une livraison au deuxième trimestre 2022. Ces nouvelles structures permettront de réguler le taux de surpopulation

économiques, il était possible, pour les notaires, d'habiliter certains de leurs clercs. Considérant que cette possibilité constituait un frein au recrutement de notaires, il a été décidé à partir du 31 décembre 2020. Pour faire face au bouleversement que cela constitue pour les clercs habilités, une passerelle a été mise en place pour permettre à ceux-ci, sous conditions d'expérience, d'acquérir la qualité de notaire et d'exercer en tant Toutefois, en Alsace et en Moselle, la situation est un peu plus compliquée. En effet, il s'y ajoute, pour les clercs habilités disposant d'une ancienneté minimale de quinze ans, l'exigence d'un concours de droit local. Les clercs en question, n'ayant eu accès à ce concours que depuis un décret du 25 juillet 2018, n'auront concrètement disposé que de deux ans pour réussir cette épreuve. Par ailleurs, outre le sacrifice que représente ce concours pour des personnes qui ont souvent à assumer des charges familiales, cette épreuve a quelque chose de dévalorisant pour des professionnels aguerris, justifiant pour certains de plus de vingt ans d'expérience,

la loi du 6 août 2015 précitée a supprimé la possibilité, pour les notaires, d'habiliter certains de leurs clercs à donner lecture des actes et des lois et à recueillir les signatures des parties. Ces dispositions étant applicables en Alsace-Moselle, les habilitations des clercs alsaciens ou mosellans prendront donc fin, comme sur le reste du territoire français, au 31 décembre 2020. Afin de compenser les effets de cette mesure, le Gouvernement, au travers de l'article 17 du décret du 20 mai 2016, permet aux clercs habilités justifiant de quinze années d'expérience d'être dispensés des conditions de diplôme pour accéder aux fonctions de notaire. L'ensemble des clercs habilités du territoire français bénéficiant des mêmes dispenses à situation égale, il ne saurait y avoir de rupture d'égalité entre les clercs alsaciens ou mosellans et les autres. L'exigence supplémentaire, pour les clercs souhaitant accéder au notariat en Alsace-Moselle, de passer le concours prévu à l'article 110 du décret du 5 juillet 1973 tient aux particularités juridiques locales,

Toutefois, l'élaboration du rapport prévu par l'article 52, paragraphe VII, de la loi du 6 août 2015, relatif à l'opportunité d'étendre en Alsace-Moselle le dispositif de liberté d'installation, pourra être l'occasion d'étudier les modalités d'assouplissement des conditions d'accès à la profession de notaire pour les clercs

d'État, permettez-moi d'insister sur le caractère singulier de la situation de ces clercs, dont certains ne souhaitent même pas devenir notaires. Sans ce concours de droit ils subiront une véritable régression de leur carrière. Ils seront déclassés. En conséquence, je vous serai extrêmement reconnaissante de bien vouloir ouvrir le dialogue avec ces professionnels, afin de dégager une solution qui leur permette d'achever sereinement leur carrière. Il n'y aura pas de solution sans dialogue.

Depuis plusieurs mois, ils lancent un cri d'alarme pour dénoncer leur suractivité et leur difficulté à compenser les carences en ambulances privées, très vite surchargées. Dans 80 % des cas, ces interventions ne nécessitent pas leur présence, puisqu'il s'agit de simple transport sanitaire. au service départemental d'incendie et de secours (SDIS), mais lui est indemnisée à un forfait fixé, au niveau national, à 121 euros. Faute d'une augmentation de moyens, les pompiers menacent de ne plus assurer ces interventions, dont le nombre a triplé en cinq ans. service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) des trajets effectués par les services d'incendie et de secours. Dans l'Aisne, les établissements sièges de SMUR et les services d'incendie et de secours ne sont toujours pas parvenus à trouver un accord financier. En l'absence de conventions signées, les établissements de santé n'ont pas honoré leurs factures et sont donc poursuivis au tribunal pour non-paiement. Vous avez affirmé ici même, le 2 juillet dernier, que l'agence régionale de santé (ARS) des Hauts-de-France travaillait activement à une solution. Pourriez-vous m'indiquer où en sont les travaux aujourd'hui ? Peut-on réellement espérer la conclusion d'un accord satisfaisant pour les deux parties ? Plus globalement, comment envisagez-vous de revaloriser la condition des sapeurs-pompiers, dont la mission est d'abord de gérer les urgences, et non de jouer aux brancardiers ?

Il s'agit alors d'une carence ambulancière, qui fait l'objet d'une indemnisation du SDIS par l'ARS sur son fonds d'intervention.

C'est la raison pour laquelle des travaux régionaux sont menés par l'ARS en lien avec les SAMU, les SDIS, mais aussi les associations des transports sanitaires urgents (ATSU) de la région. À titre d'illustration, dans l'Aisne, département particulièrement touché par l'accroissement de ces carences, sous l'égide de l'ARS et de la préfecture, ont été actées, en présence des acteurs hospitaliers, des représentants des transporteurs et du SDIS, un certain nombre d'actions et de décisions.

entre les établissements de santé et le SDIS. Les travaux se poursuivent pour arriver à un compromis indispensable à l'élaboration d'un cadre tarifaire. À plus long terme, des modifications organisationnelles substantielles pourront intervenir à la suite de la refonte en cours du référentiel du secours d'urgence à personne et de l'aide médicale urgente, du référentiel de la prise en charge ambulancière de l'urgence préhospitalière, ainsi que du cadre réglementaire de la garde ambulancière. Telles sont, madame la sénatrice, l'ensemble des actions qui sont menées, sous l'égide de l'ARS, par les différents acteurs territoriaux.

À ce jour, il n'existe aucun traitement qui permette d'en guérir, mais l'espérance de vie des patients s'allonge. Les recherches ont établi différentes stratégies de traitement des malades atteints de mucoviscidose, qui permettent, d'une part, de ralentir la progression de la maladie et ses conséquences sur l'organisme et, d'autre part, de vivre mieux avec la maladie. Ces stratégies de traitement reposent sur l'intervention pluridisciplinaire- médecins spécialistes, infirmiers de coordination, kinésithérapeutes, psychologues, diététiciens -, la mise en place de traitements symptomatiques et l'émergence de médicaments innovants. Il est à noter que, actuellement, ces médicaments sont peu nombreux et ne sont pas accessibles à l'ensemble des 7 500 personnes atteintes de la maladie. Les centres de ressources et de compétences de la mucoviscidose (CRCM) disposent d'à peine la moitié du nombre de soignants C'est ainsi que l'association Vaincre la mucoviscidose se voit contrainte de pallier l'insuffisance de financement de ces centres, en finançant, chaque année, une vingtaine de postes de soignants, pour un montant annuel de 900 000 euros environ pour les six dernières années. Cette situation, résultant de l'obligation de pallier

et subis par les malades. Je demande donc au Gouvernement s'il a l'intention de répondre aux besoins des malades atteints par la mucoviscidose en assurant aux CRCM un financement adéquat. Je précise que ma question avait été déposée avant l'examen du projet

le financement des centres de ressources et de compétences de la mucoviscidose et la mobilisation de tous autour de cette prise en charge ont permis d'accroître l'espérance de vie des patients atteints de mucoviscidose. On ne peut évidemment que s'en féliciter. Vous évoquez la question de la dotation.

» (Piramig), la mission d'intérêt général (MIG) « ne finance pas l'ensemble du fonctionnement du CRMR, mais seulement l'activité de coordination, d'animation du réseau et certains éléments des missions de recours ou expertise, notamment réalisées sans traiter nominativement d'un patient.

En 2019, grâce au troisième plan national maladies rares, ont été délégués 30 000 euros supplémentaires pour la réalisation de parcours de diagnostic uniforme, 20 000 euros pour l'acquisition d'un outil de réunions pluridisciplinaires ou encore 15 000 euros pour la rédaction de protocoles nationaux de diagnostic et de soins. Des financements supplémentaires seront délégués d'ici à décembre prochain pour la réalisation de programmes d'éducation thérapeutique du patient, mais également de formation. En outre, le financement des plateformes d'expertise- d'expertise- 2 millions d'euros en 2019 pour dix plateformes -permettra de mutualiser certaines fonctions et de redonner de la « marge » aux CRCM. Ces plateformes contribueront ainsi à améliorer le parcours du patient et à faciliter, entre autres, sa prise en charge médico-sociale. Enfin, sur les aspects organisationnels,

avec l'insuffisance de financement des postes de soignants, pour une association comme Vaincre la mucoviscidose, met en danger la qualité et la capacité de la recherche.

Au sein de son département des Bouches-du-Rhône, les populations sont particulièrement exposées à différents types de pollution, liés aux zones industrielles de l'étang de Berre et du golfe de Fos, à l'usine Alteo de Gardanne ou encore, à Marseille,

hospitalo-universitaires, de chercheurs, de juristes, d'épidémiologistes ainsi que d'élus locaux et nationaux. Ces derniers demandent, afin de mieux accompagner l'évaluation des risques sanitaires, la mise en place d'un registre des malformations congénitales et d'un registre d'un registre général des cancers sur le territoire de la métropole Aix-Marseille-Provence et sur l'ensemble du territoire national. Monsieur le secrétaire d'État, comment le Gouvernement entend-il mieux appréhender à l'avenir les problématiques liées à la santé environnementale ? La parole

permet de disposer de chiffres robustes, le dispositif national s'appuyant sur les données des 27 registres de cancers, lesquels couvrent environ 22 % de la population française métropolitaine et trois départements et régions d'outre-mer. Pour les enfants, le registre national des cancers de l'enfant est exhaustif sur l'ensemble du territoire national depuis 2011. En juin dernier, le directeur général de la santé a saisi le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) pour qu'il mène une réflexion sur les registres et sur leur place au regard des autres outils épidémiologiques disponibles. Les conclusions de cette instance seront utiles pour la définition d'un dispositif renouvelé, répondant à la préoccupation que vous avez pu exprimer. S'agissant plus spécifiquement du territoire d'Aix-Marseille-Provence-Alpes-Côte d'Azur, les résultats de l'observatoire Revela 13, porté par l'agence régionale de santé depuis 2012, avec l'appui de Santé publique France, ont été restitués en juillet dernier. Ils indiquent, pour certaines localisations, des taux d'incidence plus élevés ont été observés pour la France métropolitaine et une répartition non homogène sur le département. Seule, cette observation ne permet pas de déterminer les facteurs d'expositions qui pourraient expliquer ce constat. Elle sera donc complétée par d'autres études, en lien avec l'Institut national du cancer et Santé publique France. Vous m'avez également interrogé sur la création d'un registre national et régional des malformations congénitales. Le premier rapport du Comité d'experts scientifiques sur les agénésies transverses des membres supérieurs, daté de juillet 2019, ne recommande pas, pour la surveillance des malformations congénitales, la création d'un registre national. Les six registres actuels couvrent d'ores et déjà 19 % des naissances en France. Ils permettent ainsi une évaluation globale des principales malformations en France. Le rapport recommande, en en revanche, la création d'un septième registre dans une zone non couverte, répondant à des critères complémentaires des registres existants, en termes à la fois de populations et d'expositions à risque, notamment dans le champ environnemental. Cette action devrait être engagée très prochainement. Afin de répondre aux enjeux posés par les questions de santé, en lien avec les facteurs environnementaux, les ARS, en lien avec l'État et les régions, copilotent les plans régionaux santé environnement (PRSE). En région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le PRSE 3 est structuré autour de neuf axes thématiques : l'air, l'eau, l'habitat, le bruit, les risques émergents, le changement climatique, l'urbanisme, les déchets et l'alimentation. Il a permis le financement de plus de 90 projets. Pour conclure, ces enjeux

médicale ont vu leur système de formation profondément modifié, et ce, malheureusement, sans prise en compte de leurs revendications légitimes. Alors qu'ils demandaient une formation de deux ans, ils ont vu la durée

attirer son attention sur le fait que les assistants de régulation médicale attendent toujours une revalorisation salariale, au regard des missions essentielles qu'ils accomplissent et des responsabilités qui leur incombent.

ce nouveau dispositif suscite beaucoup d'inquiétudes et de craintes des professionnels du secteur, notamment concernant les personnes qui seraient en charge de recevoir les appels. De quelles formations ces dernières

et appliquée de manière disparate sur le territoire qui existe aujourd'hui a été jugée comme ne répondant plus aux besoins des professionnels ni aux nouveaux enjeux de la régulation médicale. Ainsi, à l'issue d'une phase de concertation engagée en 2018 avec l'ensemble des professionnels concernés, une nouvelle formation des ARM a été mise en place depuis septembre 2019. Ce nouveau dispositif consiste en une formation initiale d'une année, délivrée par des structures agréées par le ministère chargé de la santé, qui doivent satisfaire à des appels à projets exigeants. Cette nouvelle formation est désormais obligatoire avant l'entrée en fonctions des futurs ARM recrutés dans les centres 15.

En cohérence avec cette évolution, le régime indemnitaire des ARM a été revalorisé, afin de rendre compte des compétences nouvelles de cette profession. C'est ainsi qu'une prime de 120 euros bruts a été créée cet automne. Sa création a été publiée au le 5 novembre dernier, avec une effectivité sur les payes de novembre.

d'une part, en prévoyant des dérogations à la mise en accessibilité des établissements recevant du public (ERP) en cas d'impossibilité technique et, d'autre part, en posant le principe général d'accessibilité pour ces établissements. Les meublés de tourisme ne sont soumis aux obligations de sécurité et d'accessibilité des ERP qu'au-delà d'une capacité de quinze personnes. En deçà, une simple déclaration préalable à la mairie suivie de l'enregistrement auprès du greffe du tribunal de commerce suffit. L'immatriculation au registre du commerce n'est d'ailleurs obligatoire que si l'activité est exercée à titre « habituel ou principal », ce qui ne concerne qu'une infime partie des gîtes, notamment en zone rurale.

en subdivisant leur bien en plusieurs « lots » de moins de quinze personnes. Dans mon département de l'Eure, certains sites gérés par des organismes agréés par la préfecture de région au titre du programme « vacances adaptées organisées » ne sont pas accessibles aux personnes en situation de handicap. Ainsi, sur les 287 gîtes eurois référencés, une dizaine de gîtes seulement ont à respecter les règles. Il existe donc un vide réglementaire, préjudiciable aux personnes en situation de handicap. S'il paraît exagéré de restreindre trop fortement les dérogations permettant aux propriétaires de rentabiliser leur bien face à la concurrence toujours plus grande d'Airbnb, il est essentiel d'envisager un meilleur encadrement. Aussi, serait-il possible d'envisager l'extension du cadre légal prévu pour les ERP à l'ensemble des meublés de tourisme, quelle que soit leur taille, tout en assurant la vérification de leur bien-fondé par un service de contrôle spécifiquement formé

La chambre d'hôtes est définie légalement depuis la loi du 14 avril 2006 : « Les chambres d'hôtes sont des chambres meublées situées chez l'habitant en vue d'accueillir des touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations. Cette définition est complétée au niveau réglementaire : « L'activité de location de chambres d'hôtes mentionnée à l'article L. 324-3 est la fourniture groupée de la nuitée et du petit-déjeuner. Elle est limitée à un nombre maximal de cinq chambres pour une capacité maximale d'accueil de quinze personnes. L'accueil est assuré par l'habitant. » Ce seuil de quinze personnes a été fixé en cohérence avec la réglementation incendie, qui fixe le seuil d'effectif public à partir duquel l'établissement est assujetti à la réglementation des établissements recevant du public de cinquième catégorie. Les ERP sont, quant à eux, définis dans le code de la construction et de l'habitation. Ils désignent les lieux publics ou privés accueillant des clients ou des utilisateurs autres que les employés, à l'exception des chambres d'hôtes et des gîtes ayant une capacité d'accueil allant jusqu'à quinze personnes au maximum. En conséquence, les chambres d'hôtes que sont les meublés de tourisme comportant un nombre maximal de cinq chambres pour une capacité maximale d'accueil de quinze personnes dépendent de la réglementation afférente aux logements pour lesquels il n'y a obligation de mise en accessibilité que pour les constructions neuves. De ce fait, les meublés de tourisme d'une capacité maximale d'accueil de quinze personnes installés dans des bâtiments existants, sans qu'il soit réalisé de travaux soumis à permis de construire, ne sont pas concernés par l'obligation d'accessibilité. Dans ces conditions, les meublés de tourisme sont astreints aux mêmes obligations que les locations de courte durée chez le particulier. De fait, il s'agit d'une location chez un particulier. La subdivision du bâti en plusieurs « lots » de moins de quinze personnes permet parfois de contourner la réglementation. C'est un biais qu'il est difficile de contrer, mais qui n'est pas loi générale. En effet, il ressort de l'examen des 5 000 établissements labellisés « tourisme et handicap », hôtels, restaurants, musées et autres établissements divers que 50 % d'entre eux sont précisément des meublés de tourisme, ce qui atteste de la volonté de 2 500

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, en août dernier, dans le cadre d'une question écrite, j'ai tâché d'attirer l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur l'opportunité de déclarer l'alimentation « grande cause nationale 2020

au patrimoine culturel immatériel de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco). La place de l'alimentation en France est, vous le savez, intimement liée à notre histoire, à nos territoires et à son rôle social. Je me permets de souligner que, parallèlement à l'existence d'une gastronomie d'excellence, que le monde entier nous reconnaît, des familles peinent malheureusement encore à se nourrir suffisamment et correctement chaque jour. pour cette raison que, lancés par Coluche en 1985, les Restaurants du coeur viennent de reprendre leur campagne. Ils distribueront, cette année encore, 130 millions de repas. Cette aide alimentaire constitue le volet fondamental de l'aide à la personne et représente le premier pas vers la réinsertion pour les 860 000 personnes qui en sont bénéficiaires. Je veux ajouter que, dans sa déclaration de politique générale, le Premier ministre a invité la classe politique

Pour toutes ces raisons, je me permets, par votre intermédiaire, madame la secrétaire d'État, d'interroger le ministre Didier Guillaume sur l'opportunité de déclarer l'alimentation « grande cause nationale » en 2020.

Vous avez raison, nous pouvons et nous devons être fiers de notre alimentation en France. Elle est sûre, saine et durable. À l'heure où les liens n'ont jamais été aussi distendus entre agriculteurs et consommateurs, il me paraît essentiel de rappeler que notre pays est un pays d'excellence agricole et alimentaire. L'alimentation est aussi porteuse de nombreux enjeux. Parallèlement aux enjeux nutritionnels, facteurs de santé, la promotion d'une alimentation de qualité, ancrée dans les territoires, en lien avec une agriculture résiliente, tournée vers l'agroécologie pour répondre aux enjeux de la transition écologique, est une priorité pour le Gouvernement. Ainsi, une approche cohérente et interministérielle de l'action publique doit recouvrir tous les enjeux attachés à notre alimentation, en s'appuyant sur l'ensemble des acteurs et des parties prenantes de la chaîne alimentaire.

vise à répondre de façon globale et cohérente à ces enjeux avec deux plans phares : le programme national pour l'alimentation (PNA) et le programme national nutrition santé (PNNS). Ces plans déclinent des programmes d'action pour les années 2019 à 2023 afin de faire évoluer l'offre alimentaire, de lutter contre la précarité et le gaspillage alimentaires, favoriser la relocalisation de notre alimentation, mais également de renforcer l'éducation à l'alimentation et de promouvoir notre patrimoine culinaire d'exception. Ces programmes sont déclinés dans chacune des régions et des territoires français.

Dès lors, même si le label « grande cause nationale » peut être appliqué à l'alimentation au regard de son importance et des nombreux chantiers en cours, il ne semble pas nécessaire de le mettre en oeuvre, l'alimentation étant déjà au coeur des politiques portées par le Gouvernement depuis 2017.

je m'interroge sur le calcul du pourcentage de grévistes qui déclenche le service d'accueil des élèves par les municipalités. Vous n'êtes pas sans savoir les difficultés importantes auxquelles se trouvent confrontés les maires et élus de nos communes- notamment rurales -pour mettre en place l'obligation d'accueil des enfants. La loi du 20 août 2008 a en effet instauré un droit d'accueil pour les élèves pendant le temps scolaire en cas de grève des enseignants. Le code de l'éducation dispose ainsi, en son article L. 133-4 que « la commune met en place le service d'accueil à destination des élèves d'une école maternelle ou élémentaire publique située sur son territoire lorsque le nombre de personnes qui ont déclaré leur intention de participer à la grève en application du premier alinéa est égal ou supérieur à 25 % du nombre de personnes qui exercent des fonctions d'enseignement dans cette école

Les considérer uniquement s'ils ont déclaré leur intention de participer à la grève fausse la valeur du nombre total de personnes exerçant des fonctions d'enseignement dans ledit établissement et semble injuste aux yeux des communes qui doivent prendre en charge l'accueil des élèves.

Il est indispensable, madame la secrétaire d'État, de clarifier le mode de calcul du pourcentage de personnes, dans un établissement public donné, ayant déclaré leur intention de participer à une grève et ainsi de préciser quel personnel est reconnu comme « exerçant des fonctions d'enseignement

Comme vous l'avez souligné, la réglementation est claire : une commune doit mettre en place un service d'accueil à destination des élèves d'une école maternelle ou élémentaire située sur son territoire à partir du moment où 25 % du nombre de personnes qui exercent des fonctions d'enseignement dans l'école concernée ont déclaré leur intention de participer à la grève. S'agissant du périmètre des personnels à décompter, le premier alinéa de l'article L. 133-4 du code de l'éducation précise que « toute personne exerçant des fonctions d'enseignement dans une école maternelle ou élémentaire publique est soumise à une obligation de déclaration préalable de son intention de participer à une grève. Le principe est que la déclaration préalable n'est obligatoire que pour les « professeurs » dont l'absence prive les enfants du seul adulte qui les a « en charge ». Les personnes qui interviennent dans les classes en présence de l'enseignant ne doivent donc pas être comptées. En outre, pour simplifier les modes de décompte, les règles suivantes ont été retenues : le décompte se fait exclusivement par agent- l'agent à temps partiel est compté pour un un ; le professeur en service partagé est pris en compte dans chaque école dans laquelle il effectue un service d'enseignement ; les directeurs d'école disposant d'une décharge totale d'enseignement ne sont pas décomptés.

Les langues régionales jouent leur rôle dans l'enracinement qui fait la force des régions. Nous allons pérenniser leur enseignement. » Ce sont les mots du président Emmanuel Macron, qui n'a cessé d'affirmer son engagement pour l'enseignement des langues régionales à l'école. Le francoprovencal, ou savoyard, s'est mis en place sur une partie des Alpes du Nord, comprenant mon département, la Savoie, au cours du premier millénaire et perdure depuis plus de soixante générations. Cette langue a des origines essentiellement latines, avec quelques traces de celte. On compte en France, selon le CNRS, plus de 126 langues régionales, dont le francoprovencal. Ces langues sont l'histoire même de nos régions et permettent de promouvoir la diversité des territoires et des populations qui y habitent. Des groupes de locuteurs de cette langue travaillent à la sauvegarde de ce patrimoine vivant en faisant intervenir des enseignants et des bénévoles, ainsi qu'en organisant des groupes de théâtre et de chants en francoprovencal dans les écoles des départements concernés tels que la Savoie, la Haute-Savoie, l'Isère, l'Ain, le Rhône et la Loire. langue est également parlée dans une partie de la Suisse et de l'Italie. Par ailleurs, des rencontres internationales de locuteurs ont lieu chaque année. C'est d'ailleurs sur ce sujet que s'est tenue une conférence de travail le samedi 5 octobre au Sénat, avec des représentants de ces régions, mais aussi avec des représentants des associations parisiennes d'émigrés valdôtains et savoyards. Ces initiatives traduisent la volonté de ne pas voir s'éteindre cette partie de notre culture, reconnue à l'article 75-1 de la Constitution. Pourtant, les langues régionales ont été classées par l'Unesco comme « en grand danger d'extinction ». La crainte de les voir disparaître est forte en Savoie, où les élus, les professeurs et les familles souhaitent en préserver l'apprentissage. Afin de continuer de protéger et de promouvoir ces langues, il est nécessaire de les transmettre aux plus jeunes. Pour réussir cette transmission, leur enseignement doit passer par nos écoles primaires, nos collèges et nos lycées. Cependant, le francoprovençal n'est toujours pas reconnu par l'éducation nationale, malgré des demandes répétées depuis plusieurs décennies, alors que d'autres langues régionales telles que l'occitan, l'alsacien, le breton ou le créole le sont. Les Savoyards qui veulent présenter cette langue au baccalauréat sont obligés de passer une épreuve de langue occitane, ce qui n'est pas la même chose. Il est injuste qu'une telle inégalité perdure. Le francoprovençal doit pouvoir être proposé aux examens du baccalauréat. Je souhaite donc savoir, madame la secrétaire d'État, si le Gouvernement envisage d'ajouter le francoprovençal, ou savoyard, au nombre des langues régionales proposées aux épreuves du baccalauréat.

La préservation et la transmission des différentes formes du patrimoine des régions françaises- linguistique et culturel -font l'objet de la plus grande attention de la part du ministère de l'éducation nationale. C'est dans cet esprit qu'est examinée la situation du francoprovençal qui ne fait pas l'objet d'un enseignement de langue et culture régionale tel que le décrit la circulaire du 12 avril 2017. L'introduction d'un nouvel enseignement de langue vivante dans notre système scolaire, de l'école primaire au baccalauréat, doit être étudiée au regard de nombreux critères, tels que sa zone d'implantation et de diffusion, le nombre de locuteurs potentiels et le degré d'imprégnation et d'utilisation de la langue par la population, le corpus disponible dans les différents registres littéraires ... Ainsi, la situation du francoprovençal doit être appréciée avec finesse et discernement, au regard de l'ensemble de ces éléments. Le nombre restreint de locuteurs, d'enseignants, de formateurs et de spécialistes, ainsi que le manque de stabilité de la norme grammaticale de cette langue ne nous permettent pas d'envisager une inscription du francoprovençal sur la liste des langues étudiées dans notre système scolaire. Pour autant, et vous l'avez souligné, la sensibilisation au francoprovençal et à la culture qu'il porte peut faire l'objet d'activités éducatives et culturelles complémentaires conduites durant le temps périscolaire en lien, par exemple, avec des associations locales bénéficiant d'un agrément pour intervenir en milieu scolaire. Ainsi, signalons que la langue est enseignée dans l'académie de Grenoble depuis trente ans selon les modalités suivantes : une à trois heures de sensibilisation dans les établissements et écoles ; une initiation en école primaire dans le cadre de projets culturels une à deux heures dispensées en collège et lycée ; et une sensibilisation en école supérieure du professorat et de l'éducation.

Les discussions de la loi sur l'économie circulaire ont rappelé l'importance de la bioéconomie dans la réduction des déchets et dans la lutte contre les gaz à effet de serre. Vous le savez, madame la secrétaire d'État, agriculture et bioéconomie sont des atouts importants de notre pays. La Marne a, sur son territoire, l'un des plus importants pôles de compétitivité européens en matière de bioéconomie et des agriculteurs innovants, compétitifs et durables.

la loi a été promulguée voilà plus de trois ans et le décret n'est toujours pas publié. L'article 144 dispose : « La commande publique tient compte notamment de la performance environnementale des produits, en particulier de leur caractère biosourcé. Il fait de cette commande un levier de développement durable et constitue un encouragement au développement des produits biosourcés qui représentent, pour la France, des opportunités écologiques et économiques. Issus de matières renouvelables, les produits biosourcés contribuent à la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, à l'absorption du CO2 et à l'économie de ressources, tout en stimulant l'agriculture et en réduisant les importations de matières fossiles. Si le potentiel français sur ces innovations à forte valeur ajoutée est important, le taux de croissance de la filière française de bioéconomie demeure deux fois inférieur à la moyenne européenne. La stratégie nationale élaborée par le ministère de l'agriculture en 2018 rappelle la nécessité de prendre ce décret d'application : il facilitera en effet « le recours systématique aux produits biosourcés dans les administrations et les organismes publics

cette conciliation, en matière de commande publique, c'est l'achat public durable. La France compte environ 50 000 autorités adjudicatrices et 200 000 personnes exerçant une fonction d'acheteur public. En représentant près de 10 % du PIB, la commande publique constitue donc un levier majeur pour réussir la transition écologique et solidaire de notre modèle de développement. Afin de mobiliser ce levier, le droit de la commande publique fait régulièrement l'objet des adaptations nécessaires. En effet, l'été 2015 a été marqué par la transposition en droit français de la directive européenne du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics, ce qui a permis de faciliter l'intégration des dispositions environnementales dans les marchés publics. Ainsi que vous le soulignez, l'article 144 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a introduit, au sein du code de l'environnement, un nouvel article L. 228-4 ainsi rédigé La commande publique tient compte notamment de la performance environnementale des produits, en particulier de leur caractère biosourcé. » Cette disposition ne fait pas l'objet d'un renvoi à un décret d'application et sa mise en oeuvre relève ainsi directement de la responsabilité de chaque entité adjudicatrice. Dans ce cadre, l'État assume un rôle de facilitateur des acheteurs publics dans leurs démarches. Il le fait, par exemple, en animant un inter-réseau « commande publique-développement durable » qui permet aux acheteurs d'échanger les bonnes pratiques.

de la transition écologique et solidaire. Madame la secrétaire d'État, ma question porte sur la protection des oiseaux sauvages, et plus particulièrement sur le courlis cendré qui fait partie, en France, des espèces très menacées.

Or cette décision est contraire aux engagements internationaux de la France, signataire de l'accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie, dont le courlis cendré fait partie. Le Conseil d'État, saisi par la Ligue de protection des oiseaux (LPO), a d'ailleurs ordonné, le 26 août 2019, la suspension de cet arrêté pendant la saison 2019-2020, estimant que le quota autorisé de courlis devait être égal à zéro compte tenu de l'état de mauvaise conservation de l'espèce. De plus, aucune information détaillée n'est disponible pour quantifier les prélèvements effectués chaque année en France. Il est donc impossible de déterminer le niveau de prélèvement durable de l'espèce, comme le souligne le comité d'experts sur la gestion adaptative (CEGA) dans son avis relatif à l'espèce du courlis cendré, publié le 13 mai 2019. Enfin, la LPO a déposé une plainte à l'encontre de la France auprès de la Commission européenne, portant notamment sur le courlis cendré. La Commission a jugé la plainte recevable et une procédure judiciaire est en cours au regard de la directive Oiseaux de l'Union européenne. La réponse du Gouvernement était attendue pour la fin octobre 2019. Quelle que soit l'issue de cette procédure, je souhaiterais connaître les engagements pris aujourd'hui par la France sur ce sujet. Plus précisément, quelles sont les mesures que vous comptez mettre en oeuvre pour respecter les exigences écologiques, scientifiques et réglementaires qui s'imposent ?

le courlis cendré est inscrit, pour la France, à l'annexe II de la directive concernant la conservation des oiseaux sauvages. Il s'agit donc d'une espèce chassable dans notre pays au regard de cette directive. cendré fait l'objet d'un plan d'action international de l'accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie (AEWA) qui subordonne la chasse, en France, à la mise en place d'un plan international de gestion adaptative des prélèvements. Soucieuse de l'état de conservation défavorable de cette espèce, la France participe activement aux travaux du groupe de travail international sur le courlis cendré, créé en 2017 sous l'égide de l'AEWA. Une première réunion s'est ainsi tenue en septembre 2018 en Écosse. Par la suite, le 18 septembre 2019, un sous-groupe de travail sur la gestion adaptative visant à lancer le développement du plan international de gestion adaptative des prélèvements du courlis cendré avec tous les États européens de l'aire de répartition s'est réuni à Paris. Ce plan international doit être mis en place sous l'égide de l'AEWA dans un futur proche. Le principe de gestion adaptative des espèces est inscrit dans la législation française depuis la loi du 24 juillet 2019 portant création de l'Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement. Le courlis cendré fait partie des espèces prioritaires pour lesquelles cette gestion adaptative a été engagée, dès 2019. Dans ce cadre, le comité de la gestion adaptative a été saisi et la poursuite de la chasse du courlis cendré a été limitée, sur proposition du Gouvernement, pour la saison de chasse 2019-2020, à un prélèvement maximal de 6 000 individus, soit une baisse de 20 % par rapport aux prélèvements des saisons précédentes. Ce dispositif avait pour objectif de tester, en conditions de terrain, la gestion adaptative du courlis cendré au niveau national en attendant la mise en place du plan international adaptative précité. Le Conseil d'État a estimé, en référé, que les données scientifiques sous-jacentes n'étaient pas suffisantes pour justifier l'établissement d'un quota.

vous avez appelé l'attention du secrétaire d'État aux transports sur la réalisation de la ligne à grande vitesse Montpellier-Perpignan, notamment à la suite des épisodes climatiques dramatiques que nous avons connus dans les départements de l'Aude et de l'Hérault. La ligne existante qui relie Sète à Narbonne a été endommagée en plusieurs points en raison des précipitations exceptionnelles survenues mardi 22 et mercredi 23 octobre. Je peux vous assurer que SNCF Réseau met tout en oeuvre pour assurer une réouverture complète de la ligne, attendue pour le tout début du mois de décembre. Ce n'est pas ma question ! Le principe de la ligne nouvelle ne fait pas débat et ce type d'événement exceptionnel conforte sa nécessité. Je peux vous confirmer l'engagement de l'État sur l'axe ferroviaire méditerranéen, que ce soit aux côtés de l'Espagne, dans la réalisation de la liaison internationale Perpignan-Figueras, pour le projet de ligne nouvelle Montpellier-Perpignan. L'État a sécurisé l'ensemble du tracé de l'opération en renouvelant la déclaration de projet d'intérêt général en 2018. L'exposé des motifs du projet de loi d'orientation des mobilités affiche un calendrier de réalisation de cette ligne tenable à ce jour, sur les plans opérationnel et budgétaire, avec un engagement des travaux de la section Montpellier-Béziers à un horizon de dix ans et de vingt ans pour la section Béziers-Perpignan. Sur le volet Sur le volet du financement, l'État privilégie le scénario 2 du Conseil d'orientation des infrastructures. C'est sur cette base que la réalisation des infrastructures se fera et que le budget de l'Agence de financement des infrastructures Il conviendra de réunir rapidement les cofinanceurs en vue de relancer les études préalables à l'enquête publique et d'avoir un accord de principe sur le financement des études ainsi que sur les travaux de la ligne nouvelle. Cet accord devra prendre en compte une participation européenne.

La chambre régionale des comptes en a même déduit que sa mise en oeuvre « semble compromise ». Face à ce constat, la SNCF propose de basculer partiellement une partie du trafic TER en trafic routier. Les habitants de zones de montagne isolées, les Cantaliens, par exemple, sont très inquiets, car ils craignent d'être les premiers visés par ces mesures en raison de la faible densité de population de leur département et donc d'un taux de remplissage des trains ne pouvant égaler celui des périphéries des grandes métropoles.

que les conditions météorologiques sont extrêmement défavorables en hiver. Madame la secrétaire d'État, afin d'éviter une spirale du déclin, pouvez-vous nous assurer que ces zones,

c'est-à-dire notamment les liaisons à assurer, les points d'arrêt desservis, ainsi que les éventuels services routiers effectués en substitution des services ferroviaires. Ainsi, hormis la liaison quotidienne Intercités entre Clermont-Ferrand et Béziers, la desserte des gares du Cantal est essentiellement définie par la région Auvergne-Rhône-Alpes en fonction de l'analyse qu'elle fait des besoins de mobilité des habitants de cette région. L'État, en application du principe de libre administration des collectivités territoriales, n'intervient pas dans ses choix. Par ailleurs, le Gouvernement a pleinement conscience de l'importance des petites lignes ferroviaires pour assurer la desserte de nos territoires et pour la vitalité, en particulier, des zones rurales, souvent défavorisées en matière d'offre de mobilités. Or la situation de ce réseau de lignes secondaires est préoccupante. C'est pourquoi le Gouvernement a demandé au préfet François Philizot d'établir, dans un premier temps, un état des lieux de l'état de ces lignes, des niveaux de trafic et des montants d'investissements nécessaires pour les remettre en état. Cette mission est aujourd'hui entrée dans une seconde phase, le préfet François Philizot ayant entamé un nouveau cycle de discussions avec les régions, pour élaborer avec elles, ainsi qu'avec SNCF Réseau, un plan d'action.

Or, pour être correctement couverte, la Sarthe a impérativement besoin de l'implantation d'au moins 50 nouveaux pylônes, dans la plupart des cas quadri-opérateurs. Pourtant, aujourd'hui, au dire des autorités régionales et locales, il semblerait qu'une vingtaine seulement soit prévue.

dans la résolution de la déficience en couverture mobile, permette aux territoires de bénéficier d'un véritable levier de dynamisation, aux endroits mêmes qu'ils ont, en connaissance de cause, expressément identifiés. À ce titre, 7 communes ont été identifiées par le département comme présentant potentiellement une carence de couverture. Les opérateurs, après étude, ont confirmé que 9 pylônes étaient nécessaires pour la couverture de celles-ci, dont 5 quadri-opérateurs. Aucune programmation ne peut être envisagée à ce jour pour ces pylônes, compte tenu des quotas attribués au département de la Sarthe, qui sont notoirement insuffisants. Les communes concernées sont Saint-Jean-de-la-Motte, Boëssé-le-Sec, Gesnes-le-Gandelin, Gréez-sur-Roc et Saint-Ulphace ; Mont-Saint-Jean, Marçon et

Tennie et Vaas. Par ailleurs, une liste de plus de 60 communes reste à étudier pour que les opérateurs se prononcent sur le niveau de couverture des communes ayant été repérées, depuis plus de deux ans, comme ayant des carences, dans le cadre d'une étude menée par le syndicat régional Gigalis, en collaboration avec le syndicat départemental Sarthe numérique. Aussi, madame la ministre, je souhaiterais que vous nous confirmiez la volonté de l'État de garantir ce nombre de 50 nouveaux pylônes, majoritairement quadri-opérateurs, et notamment la prise en compte des sites d'ores et déjà identifiés par les opérateurs à la suite de l'étude menée à la demande de l'équipe projet sarthoise. La parole

à généraliser la couverture mobile de qualité sur l'ensemble du territoire français, donc pour l'ensemble de nos concitoyens. Cet accord prévoit notamment la mise en place d'un dispositif de couverture ciblée, dans le cadre duquel chacun des quatre opérateurs s'est engagé à couvrir 5 000 nouveaux sites. Les dotations correspondant à chaque département sont arrêtées sur la base de quatre critères la population du département, la surface du département, les territoires de montagne et le nombre de communes du département ayant fait l'objet de signalements sur la plateforme France Mobile. Ces critères objectifs ont été définis de manière collégiale, dans le cadre d'un comité de concertation France Mobile, au sein duquel sont représentées les associations de collectivités. S'agissant des Pays de la Loire, il faut souligner l'existence du cumul

La région Pays de la Loire et le département de la Sarthe se sont donc vu attribuer une dotation importante par rapport à d'autres territoires. De fait, votre département bénéficie du dispositif de couverture ciblée. Il s'est vu attribuer six sites en 2018-2019 et six sites pour l'année 2020,

engagé dans le contrat d'avenir qu'il a signé avec la région Pays de la Loire et conscient des fortes attentes de nos concitoyens.

madame le ministre. Elle est relative à l'engagement de l'État en faveur d'une gestion économe de l'espace. Quel est le rôle des maires en France ? Au-delà du service de proximité, parmi les missions les plus stimulantes qui leur sont confiées, c'est de mener, avec leur conseil, des projets de A à Z, en montant les dossiers, en rencontrant les architectes, en prévoyant les budgets et, enfin, en atteignant l'objectif visé. Cela peut être la rénovation d'une place, la construction d'une école ou l'implantation de nouvelles habitations. Qu'importe, pourvu que les enjeux soient en adéquation avec les besoins de la population. Aussi la circulaire de l'été dernier relative à l'engagement de l'État en faveur d'une gestion économe de l'espace adressée aux préfets et à toutes les administrations liées aux territoires et leur donnant pour mission de surveiller de près

Ce qu'exige cette instruction, véritable condensé de recentralisation, madame le ministre, c'est de surtout ne rien faire, de tout abandonner, de laisser les territoires se vider. C'est le gel du périmètre des communes rurales et la surdensification des centres-villes. Comme si cela allait résoudre la crise du logement ! Est-ce vraiment la ruralité que vous voulez ? Une campagne certes verdoyante, mais sans habitant ? Ainsi, le Président de la République pourra se gausser d'avoir tenu l'engagement d'une France écologique exemplaire, plus verte qu'ailleurs.

sur le monde agricole et la biodiversité, ainsi qu'en termes de coûts pour les ménages et les collectivités. Cette instruction rappelle aux préfets les différents dispositifs qu'ils peuvent utiliser en la matière, mais insiste sur le fait que cet enjeu doit être pris

Le rôle des élus est donc primordial dans la réflexion et le dialogue permanent avec les préfets. Il s'agit aussi de sensibiliser nos concitoyens aux nouvelles formes d'habitat, moins impactantes pour l'environnement.

territoriales. Madame la ministre, je souhaite attirer votre attention sur la situation kafkaïenne dans laquelle se trouvent les porteurs de programmes d'actions de prévention des inondations et à la prévention des inondations, sur le littoral. Les lourdeurs administratives découragent trop souvent les gouvernants locaux, qui se voient imposer un empilement de procédures administratives, financières ou environnementales. La révision quasi systématique des pièces obligatoires ou encore le prolongement d'études diverses engendrant la multiplication d'avenants sont autant d'éléments concourant aux ralentissements des procédures. Dès lors, les projets de restauration de digues deviennent obsolètes et leur révision entraîne une modification des dossiers d'autorisation environnementale. Je citerai notamment l'exemple en Vendée du syndicat mixte du marais poitevin bassin du Lay. Cet organisme en charge de la Gemapi a récupéré un ensemble d'ouvrages en ruine, qui nécessiteraient trois ou quatre ans d'études préalables à leur remise en état. Il se retrouve donc dans une situation très délicate, puisqu'il est dorénavant seul responsable d'ouvrages, en l'occurrence des digues, pour lesquelles la responsabilité est demeurée floue pendant près de soixante

réparer et de construire des ouvrages pour protéger les biens et les personnes. Les travaux de construction de digues viennent seulement de s'achever à l'automne 2019. Une telle lenteur malgré l'urgence s'explique par une bureaucratie centrale éloignée du risque, par des textes réglementaires qui n'ont pas été adaptés à la compétence Gemapi et aussi par une décentralisation partielle de cette compétence. Comment pouvons-nous lutter aujourd'hui contre ces blocages administratifs et répondre ainsi à la demande de simplification des services décentralisés ?

s'agit de prévoir la réalisation de travaux sur les ouvrages hydrauliques, notamment les digues. Les PAPI ont ainsi permis, depuis le début de 2011, la réalisation d'actions pour un montant estimé à 2 milliards d'euros, dont 800 millions d'euros de participation de l'État sur le Fonds de prévention des risques naturels naturels majeurs, c'est-à-dire le fonds Barnier. Ce dispositif, s'il rencontre un indéniable succès avec 170 programmes labellisés au 1 octobre 2019, fait également l'objet de demandes de simplification, comme vous l'avez dit, tant pour ce qui concerne ses délais d'instruction que ses modalités de mise en oeuvre. Afin d'accélérer et de faciliter les procédures nécessaires à la réalisation des travaux sur des ouvrages hydrauliques, le ministère de la transition écologique et solidaire et mon ministère

tant pour la phase d'instruction que pour celle de mise en oeuvre. Elle préconise notamment, pour l'instruction, un accompagnement renforcé des services de l'État, en confortant le pouvoir d'arbitrage du préfet de département qui pourrait désigner un interlocuteur unique unique porteur de PAPI, chargé de coordonner l'ensemble des interventions et des interprétations, afin que les élus n'aient qu'un seul interlocuteur. Pour ce qui concerne la mise en oeuvre, elle invite à une meilleure adéquation des moyens humains des porteurs de PAPI, avec des ambitions affichées. Afin d'améliorer les PAPI, les services de l'État sont en outre invités à renforcer le dialogue entre eux et avec les collectivités porteuses. Le Gouvernement a donc accueilli

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, en juin 2018, le département d'Ille-et-Vilaine, comme d'autres départements, a signé avec l'État un contrat financier, qui s'inscrit dans la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022. Il ouvre la faculté de retraiter un certain nombre de dépenses, dès lors qu'une évolution de leur montant est constatée. Le département est précisément concerné par cette possibilité, dans la mesure où ses dépenses en matière d'éducation sont et seront amenées à varier sensiblement. En effet, la croissance démographique générale du département progresse à un rythme annuel de plus 1,08 %, soit le double du niveau national. Quant aux plus jeunes, les 5-19 ans, entre 2013 et 2019, leur croissance s'est avérée trois fois plus importante dans le département que la moyenne établie à l'échelle de la France. Ainsi, d'ici à cinq ans, ce sont près de 1 400 collégiens supplémentaires qui sont attendus dans les établissements publics du département. du département. Cette prévision rend impérieuse la création de trois collèges et la réalisation d'extensions multiples aux établissements existants, l'augmentation annuelle des effectifs de collégiens étant supérieure à 600. Concrètement, ces investissements auront un impact financier significatif dès l'année prochaine, estimé à environ un million d'euros. En année pleine, le coût de fonctionnement de chaque nouveau collège, avec une capacité fixée entre 700 et 800 élèves, est de l'ordre de 700 000 euros, soit un effort budgétaire représentant quelque 2 millions d'euros à compter de 2021. En d'autres termes, si cette croissance démographique témoigne de la vitalité du département et se révèle une aubaine pour l'ensemble de la région, il n'en demeure pas moins qu'elle est un défi auquel la collectivité doit répondre, pour assurer au mieux la réussite de ses élèves.

Madame la sénatrice, en effet, la loi du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques fixe un taux de croissance annuelle des dépenses réelles de fonctionnement des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements à 1,2 % sur la période 2018-2022. Des critères de modulation de ce taux d'évolution ont été prévus par la loi, pour tenir compte des caractéristiques propres à chaque collectivité. Ils prennent en compte les évolutions supérieures à la moyenne pour la population, la construction de logements, le revenu par habitant, la part des habitants en quartiers relevant de la pour les dépenses réelles de fonctionnement entre 2014 et 2016. Le département d'Ille-et-Vilaine n'était éligible à aucun de ces critères, et plus particulièrement à celui qui prend en compte la problématique de l'évolution de la population de la collectivité. En effet, bien que la croissance de la population du département d'Ille-et-Vilaine s'élève à 1,08 % en moyenne par an entre 2013 et 2018, cette progression n'est pas supérieure d'au moins 0,75 point à la moyenne nationale. De même, la moyenne annuelle du nombre de logements autorisés ayant fait l'objet d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable entre 2014 et 2016 ne dépassait pas le seuil fixé par l'article 29 de la loi de programmation. Ce seuil est de 2,5 alors que la moyenne annuelle des logements autorisés sur le nombre total de logements est de 1,76 % pour le département d'Ille-et-Vilaine.

les collectivités territoriales. Une association environnementale a fait annuler partiellement un décret relatif aux unités touristiques nouvelles (UTN), spécificité de la construction en montagne, qui s'inscrivait dans le cadre global d'une réforme visant à simplifier la procédure pour obtenir des autorisations de construction. Créées dans les années 1980 pour déroger au principe de continuité des constructions, les unités touristiques nouvelles étaient un préalable à la délivrance de toute autorisation de permis de construire. Le décret du 10 mai 2017, pris en application de la loi Montagne 2 du 28 décembre 2016, dont j'étais le rapporteur visait à rénover l'ensemble de la procédure des unités touristiques nouvelles. Le décret modifiait la procédure de création et d'extension des UTN, en actant une nouvelle répartition : « UTN structurantes » planifiées par les SCOT, les schémas de cohérence territoriale, Cette réforme visait à inciter les communes de montagne dépourvues de documents d'urbanisme à s'engager dans la voie de la planification. Le texte modifiait également plusieurs seuils existants, afin d'en corriger certains, permettait d'intégrer des projets touristiques structurants pour le territoire et de déconnecter les seuils UTN des seuils retenus pour la réalisation d'une étude d'impact, ces derniers apparaissant parfois peu pertinents au regard des échelles de planification des SCOT ou des La décision du Conseil d'État précise que le décret méconnaît l'obligation pour tous les plans et programmes de procéder à une évaluation environnementale en amont. Le Conseil d'État a donc partiellement annulé le décret, qui ne soumettait pas à une évaluation environnementale les UTN créées dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale ou par un plan local d'urbanisme.

Par ailleurs, comme une évaluation environnementale s'accompagne d'une enquête publique, il faudra également l'organiser conjointement. Dans un premier temps, je souhaiterais connaître le nombre d'UTN concernées par l'annulation du décret et des autorisations préfectorales et les conséquences juridiques pour ces projets. Je demande également au Gouvernement d'indiquer ses intentions pour alléger le dispositif, conformément à l'objectif initial défendu en son temps par le ministre Emmanuel Macron. La

par une décision du 26 juin 2019, le Conseil d'État a en effet annulé le décret du 10 mai 2017 relatif aux unités touristiques nouvelles en tant qu'il ne soumet pas à évaluation environnementale la création ou l'extension d'UTN soumises à autorisation préfectorale, en l'absence de SCOT ou de PLU, dès lors qu'elles sont susceptibles d'avoir une incidence notable sur l'environnement. Le Conseil d'État a ainsi considéré que ces UTN résiduelles sont des plans-programmes au sens du droit communautaire et que le décret aurait donc dû les soumettre à une évaluation environnementale. C'est le silence du décret sur ce sujet de l'évaluation environnementale qui est annulé. le contenu de ce décret, notamment pour ce qui concerne le régime des UTN, est validé et reste totalement opérationnel. Il n'y a donc pas lieu de le modifier. Les conséquences de cette décision de justice sont les suivantes : elle implique qu'il faut compléter les textes en vigueur pour soumettre expressément les autorisations UTN résiduelles à évaluation environnementale. Toutes les instances Toutes les instances concernées seront associées, bien sûr, à ce chantier réglementaire. Cette décision implique par ailleurs, et par définition, qu'il faut soumettre les autorisations UTN à venir à évaluation environnementale- tant que tant que les textes n'ont pas été modifiés, la jurisprudence du Conseil d'État s'applique directement. Enfin, le Conseil d'État ayant retenu la méconnaissance du droit européen en la matière, l'annulation qu'il a prononcée est rétroactive, ce qui met en exergue autorisations UTN résiduelles adoptées sans évaluation environnementale. Cependant, l'exception d'illégalité résultant de l'absence d'évaluation environnementale de l'autorisation préfectorale portant création d'une UTN devenue définitive, quelle que soit sa nature juridique, ne devrait pas pouvoir être invoquée à l'occasion de la contestation d'une autorisation d'urbanisme, et l'exécution de la décision du Conseil d'État du 26 juin 2019 n'implique donc pas de rejeter d'office les demandes d'autorisation d'urbanisme si une autorisation préfectorale portant création d'une UTN devenue définitive est irrégulière pour ce motif. Les conséquences de cette décision de justice, ainsi que les moyens de sécuriser les autorisations à venir,

et du logement. Madame la ministre, j'attire votre attention sur la situation dramatique des personnes en situation de mal-logement ou vivant à la rue. Le Président de la République s'était engagé, en juillet 2017, à ce que plus personne ne dorme dehors. Deux ans plus tard, les chiffres sont encore plus alarmants que les années précédentes. Près de 240 000 personnes vivent à la rue, privées de logement, comme le montre le vingt-quatrième rapport de la Fondation Abbé Pierre. La question du logement et de l'hébergement d'urgence revêt une acuité particulière avec la progression alarmante des violences conjugales ainsi que du nombre de personnes en proie à une précarité extrême. Les associations féministes ont dénoncé le fait qu'elles n'avaient toujours aucune précision concernant le financement des 1 000 places d'hébergement d'urgence promises par le Gouvernement pour mettre à l'abri les femmes victimes de violences. L'État doit jouer son rôle et protéger nos concitoyennes et nos concitoyens en consacrant des moyens supplémentaires à la création de nouvelles places d'hébergement d'urgence

Les crédits sont donc en constante augmentation. Mais la réponse ne peut pas être uniquement budgétaire. Par conséquent, les maraudes sont également renforcées, de même que les effectifs du 115. Récemment signée, la charte pour la coordination entre les plateformes 115 et 3919

seront au nombre de 5 715 au 31 décembre 2019. Parmi les annonces du Gouvernement lors du Grenelle des violences conjugales figure en outre- vous l'avez dit -la création de 1 000 places d'hébergement et de logement temporaires supplémentaires.

Madame la ministre, comment ne pas être indigné quand 700 enfants dorment dehors chaque nuit et quand 20 000 enfants sont logés dans des conditions très précaires voire indignes, dans des hôtels d'Île-de-France ? d'Île-de-France ? Comment ne pas être indigné alors qu'une dizaine de jeunes mères sans abri ont été refoulées de l'hôpital Trousseau, où elles étaient venues chercher refuge avec leurs enfants, mercredi 27 novembre dernier ? De plus en plus de bébés naissent dans les rues : depuis le début de l'année, on en compte 146, contre 49 en 2017. La France est pourtant signataire de la convention internationale des droits de l'enfant, dont on vient de célébrer les trente Comment le Gouvernement peut-il prétendre aider les personnes à la rue sans lutter contre les expulsions locatives- on en a dénombré 36 000 en 2018 ? Vos engagements, madame la ministre, sont bien peu de chose face à cette véritable crise humanitaire. Je vous invite à mieux lire le rapport de la Fondation Abbé Pierre et à débloquer des moyens pour toutes les associations qui accompagnent les plus fragilisés et les femmes victimes de violences. La parole

Les coupes de 2017 ont considérablement affecté la qualité du service public rendu par nos consulats, déjà exsangues, à la suite de demandes récurrentes d'économies. Les augmentations budgétaires annoncées ne nous replacent toujours pas au niveau du budget de 2016, et le manque à gagner est toujours de plusieurs millions d'euros sur chaque ligne budgétaire. Le Gouvernement a lancé la réforme dite Action publique 2022, dont je soutiens complètement le concept, qui consiste non seulement à demander à l'ambassadeur de gérer les moyens de son ambassade, mais à placer celui-ci au coeur de l'organisation interministérielle de l'État dans sa projection internationale.

Autre exemple de suppression malheureuse : celle du poste de chargé des affaires sociales à l'ambassade du Brésil, dont le titulaire veille à la bonne application de la convention sur les pensions de retraite. Cette suppression posera de graves problèmes ; les retraités n'obtiennent en effet que très tardivement, voire avec une année de retard, la libération des paiements autorisés par la Caisse dit, je voudrais centrer ma question sur la dématérialisation. Il me semble que certains pensent, à tort, qu'elle peut compenser les suppressions de postes. Elle simplifie souvent la vie de nos compatriotes à l'étranger, mais ne peut être bénéfique que si elle est accompagnée de moyens humains. Votre ministère est et sera toujours un ministère de contact. Pour leurs démarches administratives, les citoyens français ont besoin d'identifier le bon interlocuteur et d'être accompagnés, non par un écran, mais par un agent formé, compétent et dont l'expérience leur apportera les réponses attendues.

qui ne supprime pas l'accueil au guichet. La possibilité de s'inscrire en ligne au registre des Français résidant à l'étranger a été utilisée par 31 % de nos compatriotes inscrits en 2018, eux pour les onze premiers mois de l'année 2019, ce qui représente autant de nouveaux inscrits au registre qui n'auraient certainement pas tous pris le temps de se déplacer ou de prendre un rendez-vous pour se faire connaître, sachant que beaucoup d'entre eux résident à plusieurs centaines de kilomètres du premier consulat.

Nous le savons : l'activité augmente dans tous nos consulats, puisqu'elle a en gros, à l'échelle du globe, doublé depuis dix ans. La dématérialisation permet aux agents de faire face à des volumes croissants La suppression de certaines étapes leur permet de se libérer de tâches fastidieuses, notamment de la gestion du papier, et de se recentrer sur ce qui fait leur véritable valeur ajoutée, en exerçant notamment une protection consulaire- vous avez parlé de l'action sociale, qui reste pour nous une priorité. Ainsi sera offert à nos En outre- je tiens à le rappeler -, nous exerçons des fonctions régaliennes ; et aucun système informatique ou d'intelligence artificielle ne prendra de décisions régaliennes. Nous aurons toujours besoin de l'expertise poussée de nos agents,

des parlementaires, de la société civile, pour qu'enfin vous reveniez sur une très mauvaise décision que votre ministère avait prise, à savoir la fermeture du consulat de France à Moncton.

des consulats généraux, que nous maintenons ouverts avec de vrais moyens- nous les préférons à une multiplication de points de contact auxquels font défaut les moyens de leur rayonnement efficace. Moncton a une histoire particulière : ce consulat avait été installé dans la ville en 1964 par le général de Gaulle pour réaffirmer nos liens avec la communauté acadienne. Comme l'a dit Jean-Yves Le Drian la semaine dernière, ce consulat sera maintenu. Cette décision s'explique par l'attachement de la France à l'Acadie et par la volonté du Gouvernement de défendre la francophonie, puisque le Nouveau-Brunswick est la seule province officiellement bilingue du Canada, en plus d'être, avec le Québec, membre à part entière de l'Organisation internationale de la francophonie. Nous jouerons depuis ce consulat un rôle essentiel dans l'intégration de Saint-Pierre-et-Miquelon dans son environnement régional- je sais que vous êtes sensible Dans le cadre de la densification de nos relations politiques et économiques avec le Canada et notamment de l'accord économique et commercial global (CETA) entre l'Union européenne et le Canada, il nous semblait important, pour notre diplomatie économique, que ce consulat soit maintenu.

Au lendemain de la diffusion de cette décision, l'émotion était à son comble dans la communauté française, mais aussi et surtout dans toute la communauté acadienne. En octobre 2018, le Président de la République affirmait pourtant aux représentants de 84 nations réunis à l'occasion du sommet de la francophonie, à Erevan, que « la francophonie sera une force dans la mondialisation » et qu'« il faudra utiliser tous les outils pour cela ». Madame la secrétaire d'État, comment la France pouvait-elle prétendre vouloir être solidaire du fait français en Amérique du Nord et, d'un même mouvement, tourner le dos aux Acadiennes et aux Acadiens en imaginant fermer ce consulat ? Le consulat général de France dans les provinces de l'Atlantique est un outil formidable de création de richesses. Son impact a été grand, en Acadie, depuis son ouverture. Sa présence a permis de confirmer le caractère privilégié des relations entre le peuple acadien et le gouvernement français et a été à l'origine, comme vous l'avez dit, du développement de plusieurs ententes de coopération entre la France et l'Acadie.

Le consulat est aussi un acteur clé dans le développement des relations triangulaires entre la France, l'Acadie et le Québec, tant sur le plan économique que sur le plan culturel. Alors qu'une vingtaine de collectivités françaises entendent renouveler leurs jumelages existants avec des communautés acadiennes ou travaillent à en faire naître de nouveaux, alors que de nouvelles perspectives d'échanges apparaissent, la pertinence de cette présence consulaire est plus qu'avérée. le flux d'immigration française dans les provinces de l'Atlantique risquerait également de décliner, au moment où chacun voudrait le voir augmenter. Les acteurs politiques, économiques, associatifs des provinces atlantiques ont donc décrété la mobilisation générale pour appeler la France à revenir sur cette décision qui aurait eu des conséquences catastrophiques et aurait été vécue comme un nouvel abandon après le tragique épisode de 1755. Prix Goncourt 1979, Antonine Maillet a pris la plume pour rappeler au Président de la République « la ferme volonté d'une communauté de poursuivre la lutte qui dure depuis quatre siècles pour garder vivant l'un des fleurons de la France doublement millénaire transplanté en Amérique

de l'agriculture et de l'alimentation. Des artisans pêcheurs du Calvados, département que je représente au Sénat, m'ont fait part de leurs vives inquiétudes quant aux conséquences de l'activité de chalutiers industriels géants, qu'il serait plus juste d'appeler « usines flottantes », qui sillonnent la Manche. Je souhaite ici être leur porte-parole. Mesurant parfois plus de 140 mètres de long et pouvant collecter 250 tonnes de poissons en une seule journée, soit l'équivalent annuel de cinq bateaux normands, ces navires-usines pillent tout, détruisent une partie des fonds marins, de la flore, de la faune, avant de recommencer ailleurs. Techniques industrielles non raisonnées, impacts écologiques catastrophiques, mise en danger des ressources et des espèces : cette pêche au large des côtes normandes est une menace pour la ressource halieutique. Tout le monde sait que la politique européenne des quotas est d'abord dictée par la préservation des espèces et de la biodiversité et par la lutte contre le gaspillage. Il est donc difficile de comprendre qu'on laisse faire de tels « ogres des mers Après le passage dans la Manche d'un « monstre de la pêche » comme le, navire néerlandais, que pensez-vous qu'il reste, madame la secrétaire d'État, pour nos artisans pêcheurs qui travaillent dur et honnêtement toute l'année et qui, eux, régulent de fait leur production ? Alors que les pêcheurs du Calvados ont su mettre en place un modèle économique pérenne et respectueux de l'environnement, il ne peut être toléré que cet équilibre vertueux, mais fragile, soit mis en danger par une telle concurrence déloyale. Dans une période où le Brexit suscite déjà beaucoup d'inquiétudes, la France doit plus que jamais défendre sa vision d'une gestion raisonnée de la pêche : une pêche artisanale, durable et responsable. Aussi, j'aimerais savoir si le Gouvernement compte agir au niveau européen pour demander une révision de la politique commune de la pêche et ainsi faire cesser toute pratique synonyme de désastre pour l'économie locale liée à la pêche et pour l'environnement, et, le cas échéant, dans quel cadre et à quelle échéance.

qui montrent qu'il y a là un enjeu à la fois territorial et stratégique. Je tiens à excuser l'absence ce matin du ministre de l'agriculture et de l'alimentation ; nous travaillons ensemble, de manière extrêmement rapprochée, pour que, à Bruxelles, dans les cadres européens, que ce soit par le biais de la filière diplomatique ou de la filière thématique de la pêche, nous puissions avancer. Nous sommes et nous restons, avec l'Union européenne, très mobilisés contre la surpêche. Tel est le sens de la politique commune de la pêche mise en place en 2013 ; tel est le sens, également, de toutes les positions qui ont été défendues par l'Union européenne au sein des organisations internationales

Nous le faisons avec les représentants des secteurs, avec les différents comités de pêche des bassins qui entourent notre pays, sur la base d'avis scientifiques robustes. Les négociations des prochaines semaines feront l'objet de consultations régulières, comme c'est le cas pour l'ensemble des négociations relatives à cette politique commune.

le fameux bateau a effectivement transité par les eaux territoriales françaises ; il a pêché dans les eaux communautaires, pas dans les eaux françaises. Il a un quota, de 2 150 tonnes ; il pêche en particulier du chinchard, et nous avons exercé, avec le Centre national de surveillance des pêches, une veille très attentive pour nous assurer qu'il respectait

! L'Union européenne a le pouvoir de modifier cette politique commune de la pêche. Il faut d'urgence des règles strictes pour éviter que cette catastrophe n'ait des conséquences irréversibles sur le secteur de la pêche, notamment dans le Calvados et en Normandie. La parole est

et de l'alimentation. Depuis 2015, la politique agricole commune (PAC) a reconnu les surfaces pastorales comme des surfaces productives. Ces surfaces correspondent à des milieux naturels et hétérogènes, ainsi qu'à une diversité de paysages- landes, estives, parcours humides -où l'herbe et les fourrages ne sont pas toujours abondants. La France, pour tenir compte de la diversité des situations, a mis en place une méthode de calcul proratisée, qui consiste à estimer la part de surface admissible à partir du taux de recouvrement d'autres éléments non admissibles, comme les roches, les éboulis et les buissons. Le règlement Omnibus a d'ailleurs confirmé, en 2018, la reconnaissance des surfaces pâturables où l'herbe et les autres fourrages herbacés ne sont pas nécessairement prédominants. Dans les Hautes-Pyrénées, les surfaces pastorales, peu productives, représentent 145 000 hectares et constituent l'essentiel des surfaces alimentaires du cheptel du département. On y compte 955 éleveurs transhumants et on estime que pour 1 hectare de surface exploité en vallée ou en zone intermédiaire, ce sont près de 3 hectares qui qui sont valorisés et entretenus en zone pastorale. Cela participe à la qualité environnementale, à la sécurité publique et à l'économie touristique. Comme sur l'ensemble du massif pyrénéen, la reconnaissance de l'éligibilité de ces surfaces constitue un enjeu majeur pour un modèle d'agriculture familiale et pastorale : elle est indispensable au maintien d'exploitations sur des espaces riches en biodiversité, où l'élevage est souvent la seule activité permettant la valorisation et la préservation de milieux ouverts. Les éleveurs et les professionnels du secteur sont aujourd'hui très inquiets de la future réforme de la PAC pour la période 2021-2027. Ils craignent une remise en cause des aides aux surfaces pastorales en raison des difficultés de contrôle de ces espaces par la Commission européenne, alors même que ces aides ont largement contribué au rééquilibrage des subventions versées au monde de l'élevage. Pouvez-vous m'indiquer, madame la secrétaire d'État, si le Gouvernement compte éviter une modification des conditions d'éligibilité des surfaces pastorales aux aides de la PAC ?

et a obtenu leur reconnaissance dans le cadre de la PAC actuelle 2014-2020. L'importance de ces zones a conduit le Gouvernement à mobiliser cette nouvelle possibilité réglementaire pour étendre la prise en compte de ces surfaces dans trente-huit départements.

et sécuriser la gestion de ces surfaces. La bonne mise en oeuvre de la réglementation est essentielle pour sécuriser juridiquement l'admissibilité de ces surfaces aux aides européennes, et promouvoir par ce biais le maintien de l'activité pastorale dans les zones concernées. Si nous travaillons collectivement- Gouvernement, organisations professionnelles

À l'heure où nos concitoyens souhaitent que l'on revienne à une agriculture traditionnelle, il est indispensable de préserver ces aides pour soutenir économiquement le pastoralisme et l'élevage extensif. Vous l'avez souligné, ces activités participent au maintien de la qualité environnementale de ces espaces et de la biodiversité associée aux pratiques pastorales.